Chacun sera attentif au respect des uns et des autres et au respect du temps. La parole est à M. François Calvet, pour le groupe Les Républicains.

Elle porte sur le devenir du réseau routier national. Le 15 mai 2018, vous confirmiez que 50 % des chaussées étaient à renouveler et qu'un pont sur dix était en mauvais état. Des experts ont chiffré le montant des investissements à 1 milliard d'euros supplémentaires par an. Dans les deux derniers budgets de l'État, le compte n'y est pas. Plus inquiétant encore, pour la première fois, les mobilités ne figurent pas dans les objectifs du nouveau contrat de plan 2021-2027. Pourtant, le réseau routier reste un enjeu stratégique pour le désenclavement et l'économie de nos départements. Dans cette négociation du contrat de plan, pouvez-vous nous confirmer que les crédits routiers n'y figureront plus ? Parallèlement, vous entamez la concertation sur le projet de loi dit Le transfert du réseau routier national aux collectivités territoriales sera-t-il l'objet de ce projet de loi, et quels crédits y affecterez-vous ?

tout d'abord, le Gouvernement a parfaitement conscience du retard accumulé dans la régénération du réseau routier national, du fait des sous-investissements chroniques de ces dernières années. C'est la raison pour laquelle il a commandé, à l'été 2017, un rapport d'audit externe, qui a confirmé la nécessité d'un budget

L'État est donc au rendez-vous de l'objectif de maintien de la sécurité des usagers, mais aussi du désenclavement des territoires qui sont chers à votre coeur. La LOM prévoit également un financement du plan de désenclavement des territoires ruraux à hauteur de 100 millions d'euros par an.

s'agissant de la décentralisation et du projet de loi « 3D », qui sera débattu au Sénat, j'ai eu l'occasion de le dire à l'Assemblée nationale : il n'y a pas de projet systématique de décentralisation des routes, même si certaines collectivités en font la demande, notamment pour des portions de routes de leur ressort. Ensuite, afin de ne pas accumuler de nouveaux retards, le Gouvernement entend agir également en prévention sur l'état des ouvrages. Il entend mettre à disposition des collectivités les préconisations qu'il prendra pour lui-même. La parole Monsieur le secrétaire d'État, en 2012, la France occupait la première place au niveau mondial pour la qualité de ses infrastructures routières ; aujourd'hui elle occupe la dix-huitième place s'agissant de la nationale 116 Perpignan-Espagne-Andorre et l'inaction sur la ligne à grande vitesse Perpignan-Montpellier sonnent le glas du milieu rural. On est bien loin des promesses du Président de la République pendant le grand débat ! La parole est à M. Loïc Hervé, pour le groupe Union Centriste. Monsieur le président, mes chers collègues, j'aimerais poser ma question à M. le Premier ministre. Monsieur le Premier ministre, la société française va mal, et, dans nos départements, nous ressentons une montée préoccupante des tensions sociales, sur fond, notamment, de réforme des retraites. Ici, l'accès des sous-traitants à un dépôt de gaz est empêché ; là, des dockers multiplient les opérations « ports morts ». Hier matin, une coupure de courant a privé 30 000 foyers d'électricité au sud de Paris et interrompu Orlyval. Depuis plusieurs mois, nos sapeurs-pompiers sont en grève pour réclamer des moyens supplémentaires, mais également pour dénoncer les violences dont ils sont l'objet. Cette semaine a commencé par des perturbations de certaines épreuves communes de contrôle continu du nouveau baccalauréat, qui suscite de vraies inquiétudes chez les enseignants et leurs élèves. En marge de ces contestations, des incidents se sont multipliés, laissant place à la violence, mais aussi à des actions nouvelles, si bien que le Président de la République lui-même a dû quitter un théâtre en cours de représentation. C'est un fait inédit. Violences de manifestants, répliques de forces de l'ordre épuisées, actions coup de poing : notre pays vit au rythme d'une immobilisation qui suscite de vives inquiétudes chez les acteurs économiques, mais aussi la lassitude et la colère de nos concitoyens. Monsieur le Premier ministre, il est temps d'apaiser ce climat, qui est l'expression de la souffrance des Français, mais dont ils sont également les principales victimes. Quelles initiatives concrètes entendez-vous prendre pour que ce climat change et que la concorde nationale revienne ?

qui prévaut en France et sur la nécessité d'apaiser, à bien des égards, les débats et l'ensemble du pays.

les réactions sociales, lorsque des réformes sont envisagées, quelles que soient d'ailleurs les majorités qui envisagent ces réformes, sont souvent vives. J'ai le souvenir, il y a quelques années, des manifestations parfois violentes qui avaient accompagné les discussions relatives à la loi dite « El Khomri » sur le travail. Nous constatons, cette fois encore, dans la perspective des discussions parlementaires qui interviendront sur le système universel de retraite, des grèves- elles sont légales, et il n'est pas question, ici, de dénier à quiconque la possibilité de faire grève -, des manifestations- de même, personne ici ne voudrait dénier à quiconque le droit de manifester. Toutefois, nous observons aussi des comportements violents, des blocages et, parfois, des actes qui, je le dis aussi simplement que je le pense, sont totalement opposés à l'esprit du service public, totalement illégaux et, en vérité, totalement inacceptables. Vous avez évoqué, monsieur le sénateur, la coupure sauvage d'électricité qui est intervenue hier et qui a privé près de 60 000 Franciliens d'un accès au réseau, interrompant des activités économiques et des transports publics.

Je veux le dire avec clarté, monsieur le sénateur : le droit de grève est légal, y compris dans les secteurs de l'énergie, et beaucoup de ceux qui y travaillent, lorsqu'ils choisissent de faire grève, s'inscrivent dans le cadre légal. À tel point que lorsque, pour les nécessités liées à la sécurité nationale, ils sont réquisitionnés, alors même qu'ils se sont déclarés grévistes, pour assurer le bon fonctionnement des installations de production ou de distribution d'électricité, ils obtempèrent à la réquisition et respectent la loi. À ceux-là,

décident d'accomplir des actions parfaitement illégales et potentiellement dangereuses, il faut dire que leur comportement n'est pas acceptable et qu'il mène directement à des sanctions. Il ne peut pas en être autrement un dernier mot, monsieur le sénateur, puisque votre question porte sur les voies permettant de revenir à une situation apaisée ou de renouer le dialogue, pour dire deux choses. D'une part, le dialogue n'a jamais été rompu. Nous discutons depuis longtemps avec les organisations syndicales, qui ont d'ailleurs toujours accepté de venir aux réunions et aux rendez-vous que nous organisions et qui ont travaillé avec nous, certaines assumant des désaccords complets sur l'objet de la réforme que nous préparons. Il est vrai que certaines refusent par principe la construction d'un système universel et que d'autres refusent par principe un système à points, mais il est des organisations syndicales, et pas les plus négligeables d'entre elles, qui pensent que, au contraire, un système universel par répartition et par points est un bon système et peut constituer à la fois un progrès social et un élément de solidité du système de pension. Nous travaillons donc avec l'ensemble des organisations syndicales dans un esprit- je le dis et je l'assume -de confiance et de respect. je crois, monsieur le sénateur, que c'est en affirmant la nécessité du respect et de la confiance et peut-être même en assumant la logique de compromis que nous sortirons de cette tension ; c'est également en appelant à la responsabilité l'ensemble de notre société, les responsables politiques, bien entendu, qui doivent, je le crois, et ils le font régulièrement, condamner la violence et les actes illégaux, et les responsables syndicaux, qui doivent, eux aussi, assumer leurs responsabilités. Au-delà de ces chacun de nos concitoyens, dans une démocratie, doit assumer ses responsabilités. Celui qui se rend coupable d'un acte illégal ou d'un acte de coupure sauvage d'électricité doit assumer ses responsabilités et ne peut pas les renvoyer à tel ou tel autre qui lui aurait demandé de le faire ou qui justifierait qu'il commette un acte illégal. Autrement dit, la solution, c'est la responsabilité individuelle, l'engagement collectif

mes chers collègues, ? Pourquoi choisir la France ? Lundi dernier, un contrat de commande d'au moins 2 milliards d'euros de navires de plaisance a été signé avec le Premier ministre entre le transporteur maritime MSC Croisières et les Chantiers de l'Atlantique. Il précédait de quelques heures l'organisation, sous ce thème, « Choose France », d'un sommet de deux cents entrepreneurs mondiaux accueillis par notre président, Emmanuel Macron, dans ce site exceptionnel et de renommée internationale, le château de Versailles. Le contrat de 2 milliards d'euros est révélateur de ce qu'est la France. En effet, MSC Croisières est une société de navigation genevoise dont le propriétaire est un entrepreneur italien, M. Aponte. Quant aux Chantiers de l'Atlantique, il s'agit du plus grand chantier naval d'Europe, concentrant un nombre incalculable de savoir-faire français. Rappelons qu'il a été construit, en 1860, par un industriel écossais, M. Scott. C'est affirmer que, de cet industriel écossais à cet entrepreneur italien, notre pays est un territoire de développement industriel. Pourtant, pendant les trente dernières années, l'industrie française a décliné lentement, mais sûrement. Aujourd'hui, la France connaît un regain d'attractivité industrielle. Quel fayot ! Les résultats sont probants : outre ce contrat, évoquons le rapport d'Ernst & Young du 13 janvier dernier, qui confirme la pole position de la France en Europe en termes d'attractivité industrielle. À long terme, six cadres dirigeants à l'étranger sur dix considèrent que l'attrait de la France a crû au cours de deux dernières années. C'est faux ! Pouvez-vous, monsieur le secrétaire d'État, nous rappeler les raisons de cette attractivité récente ? Pourquoi choisir la France ? ? La parole est

Lévrier, je vous remercie de votre question. Et je suis heureux de constater à quel point, sur l'ensemble des travées de cette assemblée, on se réjouit de ces annonces

qui créera dans les Hauts-de-France, à Dunkerque, dans une région qui en a besoin, plusieurs centaines d'emplois. Cela nous rappelle, mesdames, messieurs les sénateurs, que, aujourd'hui, ce sont plus de 2 millions de Français, dans tous les territoires, dans toutes vos circonscriptions j'imagine, qui sont employés par des entreprises étrangères. C'est pour cette raison que cette notion d'attractivité est essentielle pour tous les emplois, dans tous nos territoires. Cette attractivité, vous avez eu l'occasion de le dire, est historiquement haute. La France est probablement aujourd'hui le pays le plus attractif d'Europe, et c'est grâce à cela, que nous avons réussi aussi à faire baisser le chômage et à faire en sorte que 500 000 Français, depuis 2017, aient retrouvé un emploi. emploi. Cette attractivité, elle ne tombe pas du ciel : elle vient bien évidemment des réformes engagées par le Gouvernement depuis deux ans, ce qui est reconnu par la communauté internationale. Mais, au-delà des réformes dans le domaine fiscal, dans le domaine du marché du travail, dans le domaine des investissements technologiques, elle vient aussi de la constance de ces efforts. Monsieur le sénateur, soyez assuré que nous continuerons dans cette direction, ... Nous voilà rassurés ! ... parce que, au bout, il s'agit du combat essentiel qui nous concerne tous : celui de l'emploi.

Mais ces sujets ne doivent pas masquer d'autres problématiques, toujours d'actualité, dont l'accueil des élèves en situation de handicap. Car passer son bac relève pour certains du parcours du combattant. Pour passer son bac, il faut en effet bénéficier d'une scolarité continue, donc d'une école pleinement inclusive, et ce depuis son plus jeune âge. Or, pour fonctionner, cette école inclusive doit pouvoir s'appuyer, à côté des enseignants, sur des personnels formés, reconnus et en nombre suffisant. La réforme de 2016 a conduit à la création d'un contrat spécifique d'accompagnant d'élève en situation de handicap (AESH) et d'un diplôme dédié.

je souhaitais pour ma part vous interroger sur le remplacement des AESH en congé maladie ou en congé maternité. En effet, les inspecteurs d'académie chargés de leur recrutement ne bénéficient d'aucune marge de manoeuvre en cas d'absence de longue durée d'un AESH. D'une part, les contrats prévoient un recrutement sur trois ans et, d'autre part, l'enveloppe est utilisée dès la rentrée et en totalité pour l'accompagnement des enfants disposant d'une notification de la maison départementale des personnes Les élèves et leurs professeurs se retrouvent donc à partager l'accompagnant d'un autre élève, ou sans accompagnant du tout, sans respecter les notifications MDPH. Monsieur le ministre, vous le savez, l'éducation connaît une crise, notamment une crise des vocations. Le nombre d'inscrits aux différents concours de recrutement est en baisse régulière. Les explications sont multiples, mais, parmi elles, figurent des conditions d'exercice plus difficiles et un mal-être général. Aussi, ma question est simple : pour ces personnels AESH indispensables qui accompagnent les citoyens en devenir, pour ces enfants à qui l'on a promis l'égalité des chances, quelles sont les mesures de simplification envisagées pour une scolarité encore plus inclusive ? auprès du ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse. Monsieur le président, mesdames, messieurs les sénateurs, monsieur le sénateur Éric Gold, permettez-moi tout d'abord d'excuser l'absence de Jean-Michel Blanquer, qui se trouve aux côtés du Président de la République, en déplacement en Israël et dans les territoires palestiniens, et qui m'a chargé de vous répondre. Vous abordez la question de l'école inclusive,

en arrivant à l'école ; c'est à l'accompagnant, lors de la rentrée, d'attendre l'arrivée de la famille et de l'enfant à l'école. Toutes les mesures que nous avons prises tendent vers cet objectif. Évidemment, il y a du retard à rattraper ; évidemment, il reste encore des difficultés, parce que nous scolarisons de plus en plus d'enfants en situation de handicap, mais les choses s'améliorent. Précisément, elles s'améliorent en matière d'accompagnement. Vous avez abordé

point par point, situation par situation, mais nous avons bon espoir et nous agissons pour que, dès l'année prochaine, les choses se stabilisent dans la durée, ... Il faut conclure ! ... car c'est bien une filière professionnelle que nous avons mise en place, au service des élèves et de leurs familles. La parole

Lors du concert budgétaire de l'automne dernier, le chef d'orchestre, Bruno Le Maire, son premier violon, Gérald Darmanin, et Olivier Dussopt, à la flûte traversière, nous ont vanté les vertus d'un budget de justice fiscale et de redistribution de la richesse. Il y eut un couac cependant, lorsque l'Insee annonça que, en 2018, quelque 400 000 de nosconcitoyens avaient basculé dans la pauvreté, portant ainsi à 14,7 % le taux de personnes vivant sous le seuil de pauvreté dans notre pays, pourtant sixième puissance économique du monde. Hier, l'ONG Oxfam publiait un rapport édifiant sur les inégalités dans notre pays. On y apprend que M. Bernard Arnault, du groupe LVMH, a accru sa fortune de 41 milliards de dollars en moins d'un an. Avec cette somme, il serait possible de verser aux 67 millions de Français- bébés compris -une prime exceptionnelle de 552 euros et 7 centimes. M. Arnault gagne 11,6 euros chaque seconde. Enfin, sa fortune est évaluée à 105,5 milliards d'euros, un montant supérieur au PIB de la Croatie et de la Côte d'Ivoire. Certes, vous allez nous réinterpréter la mélodie du ruissellement,

Mesdames, messieurs les ministres, quand allez-vous, au vu de ces données, décider de changer votre musique budgétaire et fiscale ?

socialiste et républicain. Monsieur le ministre de l'intérieur, vous avez voulu, par une circulaire aux préfets, dans un quasi-secret, rendre illisibles les résultats des élections municipales de mars prochain en modifiant le nuançage politique des listes.

sera attribuée aux listes qui auraient obtenu l'investiture d'En Marche ou du Modem, mais qui aura aussi vocation à être attribuée aux listes qui seront soutenues par ces partis », y compris quand elles ne l'auraient pas demandé, ainsi qu'aux listes dissidentes, faisant ainsi exception à la règle appliquée aux autres. Après les candidats malgré eux de 2014, voilà les candidats soutenus malgré eux de 2020 ! Une belle manoeuvre, monsieur le ministre, pour gonfler artificiellement les résultats de la majorité. Nous vous demandons donc solennellement de retirer cette circulaire bien peu conforme aux valeurs démocratiques de notre République.

divers droite » ou « divers ». C'est à partir de cette réalité que nous avons travaillé, ensemble. En outre, vous avez continué, mesdames, messieurs les sénateurs, notamment en séance publique, le 15 octobre

Monsieur le ministre, vous justifiez votre manoeuvre par une demande des associations d'élus, mais à aucun moment l'une d'elles n'a mentionné un seuil de 9 000 habitants. encore, l'Association des maires de France vous demande aujourd'hui d'y renoncer et de maintenir le seuil de 1 000 habitants à partir duquel les élections se font au scrutin de liste,

Vous paniquez face à des sondages décourageants et à la multiplication des dissidences, y compris au sein du Gouvernement. Vous avez les pires difficultés à investir des candidats pour atteindre l'objectif fixé par le Président de la République des 10 000 élus locaux Vous avez délibérément choisi de nier l'existence d'une vie politique dans 8 931 communes, représentant 23,5 millions de nos concitoyens. Vous avez délibérément opté, avec cette nuance « divers centre », ... Il faut conclure ! ... pour la stratégie du coucou, cet oiseau opportuniste qui abuse des autres en pondant dans leur nid. Monsieur le ministre, il est encore temps de retirer votre circulaire ! La parole est à M. Alain Fouché, pour le groupe Les Indépendants - République et Territoires. Territoires. Monsieur le président, monsieur le ministre de l'intérieur, mes chers collègues, depuis le 20 janvier dernier, une pétition mise en ligne par des associations de consommateurs appelle les pouvoirs publics à interdire le démarchage téléphonique. Près de 200 000 personnes l'ont déjà signée. Il ne se passe pas un jour, dans ma permanence comme dans d'autres, sans que plusieurs personnes viennent se plaindre de ces démarchages incessants.

qui permet aux consommateurs de s'inscrire gratuitement sur une liste d'opposition au démarchage, est inefficace et beaucoup trop cher pour les entreprises. Dans la proposition de loi envisagée, le coût sera encore plus élevé. Se pose la question de l'efficacité de la législation et de son respect. Un effort considérable de contrôle et d'amendes a été réalisé : est-il suffisant ? Quelles mesures le Gouvernement compte-t-il prendre pour faire cesser le démarchage téléphonique abusif, tout en préservant les emplois français ?

ce sujet, celui des appels téléphoniques non désirés, répétés et effectués à tout moment de la journée, qui constituent une véritable nuisance et empoisonnent la vie de nombre de nos concitoyens, particulièrement les personnes âgées.

pour un montant total de 2,3 millions d'euros d'amendes, soit trois fois plus qu'en 2018. Par ailleurs, la DGCCRF publie régulièrement le nom des entreprises fraudeuses. Une quinzaine de décisions ont été publiées, et cela se généralisera dans les prochains mois. Nous devons également adapter nos outils, car le cadre législatif mérite d'être renforcé. C'est le sens de la proposition de loi, portée par le député Christophe Naegelen, visant à encadrer le démarchage téléphonique et à lutter contre les appels frauduleux. Le Gouvernement a soutenu plusieurs dispositions de ce texte et proposé des améliorations sur plusieurs points. Cette proposition de loi doit permettre de lutter plus efficacement contre le démarchage téléphonique en renforçant les obligations et en prévoyant des sanctions beaucoup plus dissuasives, jusqu'à 375 000 euros d'amende, avec une attention particulière portée sur le secteur de la rénovation thermique et des cas d'interdictions sectorielles. S'il faut aller plus loin, nous irons plus loin, mais je puis vous assurer de la mobilisation du Gouvernement.

Dans certains ports, pour reprendre l'expression des manifestants : « rien ne sort, rien ne rentre », et cela dure parfois depuis deux mois. C'est honteux ! La situation que suscite ce conflit est une véritable catastrophe économique pour toute la chaîne logistique. Transporteurs routiers, transitaires ou commissionnaires de transport sont les premiers touchés, mais ce ne sont pas les seuls ; certaines usines sont en mal d'approvisionnement et le secteur agricole voit ses exportations compromises. C'est inacceptable ! Les conséquences économiques vont bien au-delà des entreprises de transport. Sans les ports, il n'y a pas de commerce extérieur. Les navires se détournent vers d'autres ports européens, et les efforts mis en oeuvre pour développer les ports français se trouvent remis en cause. Comme le faisait remarquer ce matin un chef d'entreprise, on est en train d'enterrer les ports français. La situation devient difficilement tenable pour les entreprises, notamment les PME. Nous assistons à la multiplication des mises au chômage technique. Aussi, monsieur le secrétaire quelles mesures comptez-vous prendre pour venir en aide à toutes les entreprises touchées par un conflit dont elles ne sont pas parties prenantes ? Quel soutien financier concret le Gouvernement entend-il débloquer ? Ces questions, les entreprises vous les posent : elles attendent un signal fort

que sur les trafics de racks, ou encore sur les navires de croisière, qui se sont déroutés vers d'autres ports européens, pour le moment de façon temporaire, mais possiblement, demain, de manière durable. Vous l'avez dit, le mouvement social nuit gravement non seulement à l'activité économique et à l'image des ports français, mais également à l'ensemble de la filière logistique, au premier rang desquels le fret ferroviaire et le transport routier de marchandises. C'est la raison pour laquelle j'ai réuni hier au ministère, avec Agnès Pannier-Runacher, l'ensemble des acteurs et des territoires concernés, fois pour leur annoncer les dispositifs d'accompagnement à l'intention des entreprises en difficulté et pour redonner des perspectives de moyen terme aux secteurs concernés. S'agissant des mesures de court terme,

SNCF Réseau étudiera par ailleurs les modalités de soutien aux opérateurs de fret, notamment en procédant à la non-facturation des péages qui n'ont pas été utilisés. Le Gouvernement pérennise, comme vous le savez, le dispositif d'aide aux transports combinés pour la période 2019-2023, à hauteur de 27 millions d'euros Enfin, par place portuaire, un bilan économique sera évidemment dressé, afin de prendre en compte au mieux les coûts liés aux mouvements sociaux. Vous l'avez compris, le Gouvernement est mobilisé, à court terme, pour apporter tout son soutien aux entreprises en difficulté, et, à long terme, pour poursuivre les actions structurantes visant à véritablement doper les filières d'avenir de la logistique et du monde portuaire. La parole réplique. Vous l'avez compris, il y a urgence ! Les ports sont les poumons économiques de notre pays. Il faudra redonner confiance dans les ports français. Dans certaines places portuaires, les entreprises ont perdu jusqu'à 40 % de leur chiffre d'affaires. Des mesures exceptionnelles s'imposent pour les entreprises touchées, qui sont les victimes collatérales du conflit actuel. Il ne faut pas les laisser tomber ; elles ne font que subir une situation à laquelle elles ne sont pour rien.

Madame la garde des sceaux, ministre de la justice, la question que je vous pose est liée à ce que nous vivons tous actuellement lorsque nous assistons aux audiences solennelles de rentrée des juridictions : les avocats jettent leur robe ; ils sont inquiets ; ils sont en grève.

Les avocats sont essentiels à la justice, c'est la raison pour laquelle je les rencontre très fréquemment, au niveau national comme à l'échelon local, chaque fois que je me déplace dans les différentes juridictions.

Très concrètement, depuis cette semaine, je me félicite que le Conseil national des barreaux (CNB) ait accepté de participer avec la Chancellerie à des réunions techniques ; celles-ci sont en cours au moment où je vous parle. Le Premier ministre et moi-même aurons l'occasion de rencontrer les avocats demain soir, à l'issue de ces réunions techniques, avec évidemment pour préoccupation la prise en compte de la spécificité du régime des avocats dans le cadre du régime universel. Je suis persuadée que nous arriverons à des solutions qui seront satisfaisantes pour chacun. J'aborderai tout de même un dernier point, monsieur le sénateur : bien entendu, le droit de grève est un droit constitutionnel qui, en tant que tel, doit être respecté ; je regrette toutefois que celui-ci conduise parfois à des actions de blocage,

Madame la garde des sceaux, le jour où vous aurez réussi la paupérisation complète de la profession, à l'exception des avocats d'affaires qui gagnent bien leur vie, vous

car nous sommes très nombreux à nous interroger sur cette nouvelle fantaisie suggérée par le Gouvernement au travers de la circulaire sur le « nuançage », signée de votre main. Depuis bientôt trois ans, vous nous affirmez que vos préoccupations principales sont la clarté et la transparence, et voilà que vous décrétez, sans aucune consultation, que seuls les résultats des communes de plus de 9 000 habitants seront pris en compte dans les résultats nationaux par parti, excluant ainsi du calcul 96 % des communes françaises et 54 % des électeurs. Gommer d'un trait 54 % d'un résultat pour un calcul final, il me semble que, en France, cela ne s'est jamais vu ! Cerise sur le gâteau, vous créez une nouvelle nuance, dite « divers centre », qui intégrera toute liste soutenue par La République En Marche, l'UDI et le Modem, même si la tête de liste est investie par un autre parti. C'est incroyable ! Ainsi, vous modifiez la réalité du terrain et camouflez la réelle identité des listes. Devant de telles incohérences, pourriez-vous, cette fois, nous apporter des réponses claires et précises pour justifier la pertinence de cette nouvelle circulaire ?

municipale, depuis la III République, il est d'usage de demander aux préfets d'attribuer une " nuance " aux différentes listes ». Voilà la réalité de cette « nouvelle fantaisie

Cet amendement vise à respecter [ ...] la protection de la liberté individuelle et de la liberté du choix politique. Au nom de ces deux libertés, la préfecture ne peut pas affecter une couleur politique à une liste, sans que cette liste l'ait déclarée. » M. le député

dérive dans la vie politique de notre pays. Il est insupportable pour des maires ruraux d'être classés politiquement, alors qu'ils ne le souhaitent pas. » Voilà la réponse que nous avons souhaité aborder, et, je le redis,

comprendrez, monsieur le ministre, que je ne puisse adhérer à ces explications alambiquées. Bien sûr, je sais que de nombreuses communes rurales souhaitent se présenter sans étiquette, ce que je comprends et partage totalement. Un peu de liberté nous ferait tellement de bien de là à occulter le résultat de 96 % des communes qui font la France ... C'est un comble : c'est comme si on les rayait de la carte ! Pourtant, depuis des mois, les communes essaient de vous dire de ne pas les oublier. Vous faites comme pour de nombreux sujets : de belles paroles et de belles promesses qui s'évaporent dans la nature dès que vous avez refermé votre porte. C'est peut-être pour cela que la Terre et nos océans sont si pollués, contaminés de promesses non tenues ! Sachez bien, monsieur le ministre, que nous, nous comptons avec nos communes rurales et nos territoires unis ! La parole

Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, ma question porte sur la mise en oeuvre, depuis le 1 janvier, du « reste à charge zéro », ou RAC 0, pour certaines prothèses dentaires, lunettes et prothèses auditives. Pour les lunettes, le remboursement des montures est de 100 euros maximum. On peut le vérifier désormais chez les opticiens, les produits RAC 0 ne sont pas fabriqués dans l'Hexagone. C'est un coup dur pour la filière de la lunette française. Si les marques haut de gamme s'en sortent pour le moment, les lunetiers positionnés sur le créneau inférieur fabriquer les montures dans des pays à bas coût, comme la Chine. Cette filière, dont certaines entreprises se délocalisent, a perdu près d'un tiers de ses emplois. Outre cette difficulté, les opticiens, par la diminution du remboursement des frais d'optique, craignent de subir un impact important sur leur chiffre d'affaires. C'est la même problématique pour les prothèses dentaires, dont la part fabriquée en France est réduite à la portion congrue. Quant aux cabinets dentaires, leur équilibre économique est aussi fragilisé ; les alertes sont nombreuses sur des arrêts d'activité- pour les soins courants, j'entends. Enfin, concernant les prothèses auditives, même question sur le modèle économique de leur fabrication. En outre, s'y ajoutent des interrogations quant aux performances du matériel, dont on sait qu'il est très coûteux pour les cas complexes d'hypoacousie, donc qu'il n'est pas prévu dans ce cadre. On le voit bien, madame la ministre, si la mesure RAC 0 est séduisante et décrite comme un meilleur accès aux soins, elle a aussi des conséquences négatives sur les entreprises, mais aussi sur le maintien des professionnels l'optique, de l'audition et des soins dentaires dans les territoires. J'ajouterai que, en pleine opération pour valoriser le « produire français », la disparition possible de ces savoir-faire industriels est pour le moins contradictoire. Madame la ministre, ces conséquences étaient prévisibles. Nous avions déjà alerté, au Sénat, sur ce sujet. Quelles mesures envisagez-vous pour enrayer les conséquences économiques de la mesure RAC 0 ?

La réforme du 100 % santé a été élaborée et coconstruite avec les professionnels des filières et les organismes complémentaires. Depuis le 1 janvier, elle se met en oeuvre, notamment pour les lunettes, avec des équipements sur prescription médicale totalement remboursés. Les équipements de l'offre 100 % santé sont de très grande qualité. Les montures doivent être conformes à une norme garantissant un niveau de qualité et de sécurité et disposer d'un marquage CE. Les verres ont tous été contrôlés, afin de garantir leur conformité à de hautes exigences techniques. Il a été vérifié que tous les verres sont amincis,

de tailles, de couleurs, de matières, et de la qualité. Pour vous en rendre compte, madame la sénatrice, j'ai apporté une monture du 100 % santé à 30 euros, qui est de qualité.

Madame la ministre, bien évidemment, je ne mets pas en doute vos efforts pour garantir la qualité. Ma question portait sur l'origine de fabrication des produits, qui est un réel sujet.

et solidaire, après Bordeaux, Nantes, Lyon, Perpignan, Agen et Marseille, une nouvelle coupure géante d'électricité a touché hier le Val-de-Marne. Là encore, cette coupure a été revendiquée par la CGT Énergie comme une action coup de poing contre le Gouvernement. Encore une fois, ce sont les Français qui sont affectés : 135 000 habitants privés d'électricité et de chauffage toute la matinée, dix villes touchées, ainsi que l'aéroport d'Orly et le marché de Rungis. Les feux tricolores à l'arrêt ont provoqué des accidents, et les pompiers ont dû intervenir en urgence. Les passagers du tram et d'Orlyval ont été bloqués. Pis, des personnes sont restées prisonnières dans les ascenseurs. Cela ne se passe pas dans un pays lointain où l'ordre public serait absent, mais dans le Val-de-Marne, un département de 1,4 million d'habitants qui touche notre capitale ! Il est surréaliste qu'une poignée d'individus commette en toute impunité des actes aussi dangereux, pour annoncer ensuite publiquement et tranquillement dans les médias que de nouvelles coupures vont intervenir ! Monsieur le Premier ministre, vous venez de parler d'actes illégaux inacceptables et de sanctions,

Je vous le demande simplement : que comptez-vous faire concrètement contre les responsables de ces coupures qui mettent en danger la vie des Français, et pour faire respecter le droit dans un État où, actuellement, chacun se croit tout permis croit tout permis ? La parole est à Mme la ministre de la transition écologique et solidaire. Monsieur le président, mesdames, messieurs les sénateurs, madame la sénatrice Procaccia, effectivement, une coupure sauvage a été opérée sur notre réseau électrique, hier matin, au poste Enedis de Rungis. Ce sont plus de 60 000 clients- foyers, entreprises, services publics -qui ont été affectés par cette coupure, essentiellement dans le Val-de-Marne, mais aussi dans les Hauts-de-Seine et en Essonne. Cet acte a été revendiqué par la CGT Énergie, qui nous dit pratiquer des coupures ciblées. Je pose la question : ciblées sur qui, sur quoi ? Sur les milliers de salariés du marché de Rungis, sur l'hôpital de jour d'Orly, sur une caserne de pompiers, sur les transports en commun, donc sur des milliers de foyers ... Clairement, il s'agit de coupures aveugles, qui sont très pénalisantes

la grande majorité des grévistes appliquant la loi, y compris pour assurer la sécurité de notre réseau électrique. Mais je condamne très fermement ces coupures, qui sont des actes illégaux et qui feront donc l'objet de poursuites judiciaires, puisque Enedis a déposé plainte. On peut ne pas être d'accord avec une réforme, mais nous sommes en démocratie. Il y a des cadres pour exprimer ses désaccords, au moment des élections. On peut faire grève ou manifester, mais ces coupures, comme les envahissements ou les blocages, sont clairement condamnables et feront l'objet de poursuites et de sanctions. Madame la ministre, je vous demandais quelles sanctions vous comptiez appliquer. Vous ne me parlez d'aucunes ! Vous condamnez, mais condamner ne suffit pas. L'État doit systématiquement se constituer partie civile pour chaque plainte déposée par Enedis, que vous avez cité, et par d'autres en cas de coupure de courant et, à chaque fois, demander la réparation intégrale. Parler ne suffit pas, condamner ne suffit pas, agissez, s'il vous plaît

des lieux symboliques de la République qui devraient pourtant être sanctuarisés. Vendredi dernier, c'était au collège Alain-Fournier à Orléans. Lundi, c'était dans les collèges Gérard-Philipe à Clermont-Ferrand et Paul-Jean-Louis à Saint-Laurent-du-Maroni en Guyane.

Si l'on ajoute les agissements se déroulant aux abords des établissements, il est évident que la violence scolaire est un phénomène de société contre lequel il est urgent d'agir. Or nos enseignants, dont le travail doit être salué,

Mais, sur le long terme, ces faits montrent surtout l'ampleur du travail à mener pour transmettre à notre jeunesse, c'est-à-dire les citoyens en devenir, les valeurs de tolérance, de civisme et de laïcité, qui sont inhérentes à la République. Ces valeurs se déclinent en droits et en devoirs,

l'instruction civique. Près de quatre ans plus tard, et comme le craignaient les syndicats de professeurs, il semble bien que nos enseignants ne soient pas encore suffisamment formés pour dispenser cette matière, alors que les enjeux pour notre société deviennent de plus en plus patents. Mes deux questions sont donc simples. Quel bilan tire le Gouvernement de la mise en place de l'EMC ? Plus généralement, comment compte-t-il donner à nos enseignants les moyens de transmettre efficacement les valeurs qui font vivre notre République ?

La protection de l'enfance craque. Nous ne parvenons plus à mettre correctement à l'abri ni à protéger tous les enfants qui nous sont confiés. Les structures sont saturées, et les personnels sont en grande difficulté.

À mon sens, les départements sont aujourd'hui mûrs pour se mettre autour de la table et discuter des conditions dans lesquelles les responsabilités et les moyens doivent être plus justement et plus efficacement répartis entre l'État et eux. C'est

voilà trois jours, un autre documentaire nous a tous bouleversés. Votre réponse n'est pas à la hauteur de la protection de l'enfance. Je connais votre engagement. Je sais votre envie de bien faire. Je ne voudrais pas que le documentaire de 2021 vous mette trop en difficulté.

Dans ce second cas, il peut s'agir de communes qui ne finançaient pas du tout de maternelles privées avant l'abaissement de l'âge de l'instruction obligatoire ou bien de communes qui en finançaient déjà volontairement, soit les deux tiers d'entre elles. La Haute Assemblée s'était prononcée pour une prise en charge totale des frais engagés par les communes, qu'elles aient participé ou non à la scolarisation des enfants de moins de 3 ans auparavant, cette compensation garantissant seule une égalité entre elles. L'objectif était d'assurer une mesure de justice entre communes. M. le ministre semble aller dans ce sens de l'équité entre les communes, puisqu'il a déclaré lors du débat sur la loi de finances pour 2020 que les communes recevraient une compensation en cas de hausse des dépenses obligatoires pour les écoles maternelles et élémentaires et que « personne ne perdrait d'argent dans la nouvelle configuration La parution d'un décret et d'un arrêté le 30 décembre dernier mérite un éclairage, car elle ne semble pas avoir totalement dissipé les interrogations et les craintes des élus sur le sujet. Qu'en est-il exactement ?

Albéric de Montgolfier désirait s'abstenir, Philippe Dominati souhaitait voter contre et Céline Boulay-Espéronnier désirait voter pour. Acte

est ainsi libellé : La parole est à Mme Michelle Meunier. Cet amendement vise à permettre au membre survivant du couple, s'il s'agit d'une personne pouvant porter un enfant, de poursuivre le projet parental, comme l'ont successivement recommandé l'Agence de la biomédecine, le Conseil d'État et le rapport d'information de la mission parlementaire. assistée (PMA) aux femmes seules, comme nous l'avons fait hier, et refuser à une veuve de poursuivre son projet ? Ne serait-il pas traumatisant de demander à une femme endeuillée de donner ou de détruire les embryons conçus avec son compagnon tout tout en lui proposant de poursuivre son parcours avec un tiers donneur ? Cela dit, plusieurs délais sont possibles. La loi espagnole limite le transfert à une période de six mois suivant le décès.

Notre amendement s'appuie sur la législation belge. Son adoption permettrait à la femme veuve de faire son deuil en lui laissant deux ans pour décider si, oui ou non, elle souhaite aller au terme de la PMA entamée avec son compagnon décédé, détruire les embryons ou les donner à un couple ayant besoin d'un double don.

toutes les propositions formulées s'articulent autour de la mise en place d'un délai au cours duquel le membre survivant du couple pourra exécuter la procédure de PMA qu'il avait entamée.

exécutoire seulement dans un laps de temps défini. En effet, le deuil a son rythme intrinsèque : de six mois chez certains, il est de dix ans chez d'autres. Chacun devrait avoir le droit de vivre la perte d'un être cher comme il l'entend, sans restriction dans le temps. Rien ne devrait entraver la poursuite du projet familial si l'un des parents venait à décéder avant la procédure de PMA, si ce n'est peut-être la conservation médicale des gamètes et embryons, ou encore la capacité à procréer du membre survivant du couple. Dans le droit actuel, où la procréation médicalement assistée après le décès d'un des conjoints est prohibée, les seules options ouvertes au membre survivant du couple sont soit la destruction des gamètes et embryons, soit la possibilité de les donner à un autre couple souhaitant bénéficier d'une PMA. Ajouté à la peine suscitée par la perte du conjoint, ce choix lourd de conséquences est tout simplement insurmontable pour nombre de personnes endeuillées. Il est donc nécessaire que le législateur ouvre une voie nouvelle pour

Comme certains de mes collègues l'ont précédemment mentionné, dès lors que le texte permet aux femmes seules d'avoir recours à l'AMP (assistance médicale à la procréation) avec tiers donneur, il semble délicat de trancher en faveur d'une interdiction de l'AMP. Dans une telle configuration, une une femme veuve pourrait en effet procréer en recourant aux gamètes d'un tiers donneur, mais pas à l'embryon fécondé dans le cadre du projet parental entrepris avec son conjoint décédé. Dans le même temps, il paraît essentiel, dans l'intérêt de l'enfant, d'encadrer cette pratique, afin qu'elle ne porte pas le sceau du deuil. L'amendement de Catherine Procaccia tend à rendre possible l'AMP dans un délai de six à dix-huit mois après le décès du conjoint.

le délai limite pour recourir à l'AMP, afin d'offrir toutes les conditions d'une prise de décision éclairée. Si ce sous-amendement était adopté, je voterais l'amendement de Catherine Procaccia

Actuellement, les dispositions en vigueur n'autorisent pas l'insémination en cas de décès du conjoint. Or le présent projet de loi étend la PMA aux femmes seules et aux couples de femmes. Cela signifie qu'une femme dont l'époux est décédé au cours d'un projet parental

mais bien celle de savoir si le décès d'un parent avant la naissance de l'enfant constitue un obstacle absolu au développement harmonieux de ce dernier, et donc à son intérêt supérieur. Sincèrement, je ne le crois pas. Ces enfants sont le fruit d'une volonté conjointe et d'un amour parental affirmé. Les signataires de cet amendement considèrent que la qualité de l'accueil d'un enfant venu au monde prime la conformité de sa famille. Nous pensons que la conviction d'une femme dans la solidité du projet parental qui la liait avec son époux disparu peut suffire à nourrir affectivement l'enfant qui en sera issu. issu. Il convient enfin de souligner que la rédaction de notre amendement est particulièrement prudente, puisqu'elle s'articule autour de la notion de consentement de l'époux, lequel serait recueilli et révocable. Cet amendement permet également que le projet parental se poursuive dans un délai encadré et raisonnable, compris entre six

l'ouverture de l'assistance médicale à la procréation pour les mères célibataires pourrait être acquise, je considère légitime de l'étendre également aux veuves, à

couple s'ajoutera, si la femme le souhaite, l'obligation d'engager un nouveau parcours avec un tiers donneur, alors qu'elle dispose des gamètes de son conjoint décédé ou des embryons. Cet amendement tend donc à autoriser la procréation dans des conditions d'encadrement équilibrées. serait possible lorsque l'autre membre du couple a consenti préalablement à l'insémination ou au transfert d'embryons. La naissance d'un ou de plusieurs enfants à la suite d'une insémination

désormais accueillir un autre embryon ou d'autres gamètes, dès lors que les femmes seules peuvent bénéficier d'une procédure d'assistance médicale à la procréation. Mais en aucun cas elle ne pourrait avoir recours à l'embryon qu'elle a conçu avec son défunt époux.

l'embryon n'est pas le stade ultime de l'AMP. Le fait d'avoir des embryons ou des gamètes congelés ne correspond pas à des stades successifs de la démarche d'AMP. Il ne reflète que le type d'infertilité.

pour hériter, il faut exister au moment de l'ouverture de la succession. Il faudrait donc modifier l'article 725 dudit code pour inclure, parmi les héritiers, l'enfant à naître,

consiste non pasà faire sienne l'émotion sincère et profonde exprimée par certaines femmes qui sont encore sous le choc d'un deuil extrêmement cruel, mais au contraire à prendre en compte leur souffrance et à rechercher la meilleure solution

me placer délibérément du point de vue de la femme, et non de la femme en deuil. Pour moi, il ne s'agit pas de compassion et, s'il s'agissait d'entretenir éternellement le deuil, je trouverais aussi qu'il y a quelque chose de morbide, voire de toxique.

que des femmes exportent leurs gamètes pour pouvoir procéder à l'insémination à l'étranger, là où c'est autorisé. Mes chers collègues,

Il m'a dit qu'il était dur de dire « non ». Il est dur de dire « non » à une femme qui vient de perdre son mari,

Nous débattons pour savoir si le législateur doit prendre la responsabilité d'institutionnaliser et d'encadrer la PMA qui permettrait de faire naître des enfants issus d'un père mort depuis six mois,

Respectons-nous vraiment le droit de l'enfant ? Quelles seront les répercussions psychologiques sur l'enfant ? À titre personnel, je pense qu'elles seront dramatiques. Le rôle du législateur est non pas de concrétiser les désirs des parents, mais de protéger les plus vulnérables, en l'espèce les enfants. Pour moi, politique doit rimer avec justice et il faut faire justice aux adultes et aux enfants, davantage aux enfants en raison de leur intérêt supérieur. Le législateur prendrait un risque vertigineux en encadrant de quelque manière que ce soit la PMA. Je voterai donc contre ces amendements.

mais également aux parents de la personne disparue, ce qui m'a ramené au roman populaire de Pagnol décrivant la détresse de parents ayant perdu leur fils unique. Mais ce qui m'a déterminé, c'est la liberté.

Cela m'a d'ailleurs rappelé une citation d'Oscar Wilde : « Je déteste les discussions ; elles vous font parfois changer d'avis. » Il s'agit d'un domaine éminemment compliqué.

du conjoint a été explicitement recueilli, sans quoi il y aurait un abus de pouvoir sur une personne décédée. Enfin, je me garderai de tout jugement aussi subjectif que définitif sur ce qu'est une bonne famille pour un enfant. Je ne sais pas s'il vaut mieux avoir un papa mort, un papa disparu ou évaporé, un papa inconnu, une maman, deux mamans, deux papas, un papa et une maman, avec un beau-père et une belle-mère. Je crois à la résilience et je suis convaincue que la seule chose qui compte, c'est la sécurité que l'on donne à un enfant. Et cette sécurité, on peut la garantir indépendamment des formes de famille auxquelles on se réfère. C'est pourquoi je voterai l'amendement de Catherine Procaccia.

Chacun parle avec son expérience personnelle et avec le plus grand respect pour les différentes situations dans lesquelles peuvent se trouver les couples ou les personnes isolées. Malgré tout, si l'on croit à la vie, on se résout à la mort, qui signe un coup d'arrêt à la vie. C'est la raison pour laquelle,

on ne peut que comprendre que ces femmes, dans la souffrance qui est la leur, aient envie de mener à son terme le projet qu'elles avaient élaboré avec leur conjoint. Hier, dans les arguments que j'ai opposés à la PMA pour toutes, j'ai évoqué un glissement potentiel vers la GPA. C'est mon intime conviction.

la liberté de faire. Ce n'est pas une obligation ; c'est une liberté, un choix, une possibilité. Je suis intimement persuadé que cette faculté de poursuivre

des glissements ou des dérives qui vont rendre les plus vulnérables dans l'incapacité de résister à un mouvement. Et nous verrons,

Lorsque l'on évoque les cas individuels, on ne peut qu'être en faveur de cette liberté offerte, on ne peut que respecter ce choix, cette autonomie, qui a été relevée, notamment par Mme Rossignol.

sur les incidences que l'adoption de la PMA devrait nécessairement entraîner du point de vue juridique. Il faudra forcément modifier les règles d'établissement de la filiation

En effet, vous souhaitez introduire une clause de conscience spécifique pour les professionnels de santé participant à la réalisation d'une assistance médicale à la procréation pour les couples de femmes ou des femmes non mariées.

La clause de conscience en matière d'IVG concerne l'acte d'IVG et elle oblige le médecin à réorienter les patientes vers un autre collègue. En revanche, elle ne peut en aucun cas être invoquée pour différencier des personnes qui se présentent devant un médecin.

de créer une clause de conscience spécifique à l'AMP qui ciblerait certains publics, étant rappelé que l'article 7 du code de déontologie médicale prohibe toute discrimination. » Votre proposition s'apparenterait donc à de la discrimination. concerne les autres professions de santé et tous les auxiliaires médicaux, leur situation les place dans une posture d'exécuter des actes, activité à laquelle ils ne peuvent pas se soustraire. Ils ne peuvent pas justifier d'une clause de conscience spécifique au regard de leurs fonctions. médicale à la procréation, les professionnels qui exercent au sein des services spécialisés le font en toute connaissance de cause, autour d'une activité orientée vers l'aide à la procréation. Par conséquent, une telle clause ne viserait pas à offrir la possibilité de refuser de pratiquer

que quand vous interprétez les raisonnements du Conseil d'État. Peut-être est-ce parce que votre fibre médicale vous fait aborder les questions d'humanité avec pertinence

D'ailleurs, dans les discussions au Sénat, des différences seront faites entre l'assistance médicale à la procréation pour traiter un problème d'infertilité- donc un problème médical -et l'assistance médicale à la procréation

ne veut pas mettre en oeuvre. Il y a une jurisprudence très abondante de la juridiction ordinale sous le contrôle en cassation du Conseil d'État qui définit l'étendue

L'amendement présenté par M. Retailleau est donc nécessaire si l'on veut couvrir la possibilité pour un médecin hospitalier de ne pas concourir, à l'intérieur de son service de gynécologie obstétrique, à des actes d'assistance médicale à la procréation qui n'ont pas

La FIV-ROPA n'est ni un don d'ovocytes ni une gestation pour autrui ; c'est simplement une maternité partagée au sein d'un couple de femmes.

Grâce à cette technique, que nous souhaitons inscrire dans ce projet de loi, les couples de femmes souhaitant partager la maternité et vivre activement ce processus reproductif peuvent le faire. Cela peut être motivé par un choix personnel, mais aussi par des raisons médicales,

M. Sébastien Meurant. L'article 16-8 du code civil dispose que le don des éléments du corps doit être anonyme : « Aucune information permettant d'identifier à la fois celui qui a fait don d'un élément ou d'un produit de son corps et celui qui l'a reçu ne peut être divulguée. Le donneur ne peut connaître l'identité du receveur ni le receveur celle du donneur. « En cas de nécessité thérapeutique, seuls les médecins du donneur et du receveur peuvent avoir accès aux informations permettant l'identification de ceux-ci. » La pratique qui consisterait pour une femme à accueillir un ovocyte de sa compagne reviendrait donc à contourner cette interdiction.

Dans un couple de femmes, il suffira, dans la grande majorité des cas, de pratiquer une insémination artificielle pour aboutir à une grossesse. La femme qui portera l'enfant ne subira pas de stimulation ovarienne ; on lui inséminera simplement dans l'utérus

Nous sommes sensibles à la volonté de deux mères de participer au projet parental, mais cette conception de la double maternité entre en réalité en contradiction avec toute la philosophie de ce projet de loi, notamment avec l'ouverture de l'AMP aux couples de femmes.

sont ceux qui élèvent l'enfant et lui apportent amour et sécurité. Pour cette raison, le Gouvernement est défavorable aux amendements défendus par Mmes Meunier et Cohen. Quant à l'amendement de M. Meurant, il est déjà satisfait ; j'en propose donc le retrait.

Cet amendement vise à maintenir l'interdiction du double don, afin de conserver ce lien biologique avec au moins l'un des deux parents. Nous considérons en effet que cette évolution n'est pas un progrès pour l'enfant.

L'enfant qui en serait issu ne partagerait donc aucun patrimoine génétique avec ses parents. Cette disposition, en plus de priver un enfant de ses parents biologiques, risquerait d'ouvrir la porte, demain, à un marché de la procréation en permettant aux parents de choisir les caractéristiques génétiques de leur enfant.

été favorables à la levée de l'interdiction du double don de gamètes ; elles faisaient justement valoir que l'embryon donné par un couple qui n'a plus de projet parental hérite tout de même d'une histoire, alors que l'embryon issu d'un double don de gamètes commence son histoire avec le ou les parents qui souhaitent

l'impression qu'on essaie de revenir en arrière vers une conception de la famille qui est largement dépassée. Avant 1972, année qui a vu une importante réforme de la filiation- ce n'est pas si vieux ! -,

peut-être encore théologique, mais en tout cas largement dépassée. Alors, parler aujourd'hui de lignée dans le cas de la PMA me paraît extrêmement rétrograde J'apprécie la leçon d'histoire que vient de nous donner Jacques Bigot, mais je voudrais revenir à la discussion présente. La question des origines génétiques d'une personne née d'une assistance médicale à la procréation avec donneur va nous occuper encore assez longuement pendant nos débats.

on provoque une grossesse avec un embryon qui est génétiquement étranger à la mère comme au père. L'enfant n'aura plus aucun lien génétique avec les parents qui vont l'élever.

actuelle n'est pas le résultat de processus qui se dérouleraient sans encadrement médical, sans raison ni motivation.